l'amendement n° 163 rectifié. L'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 a prévu le financement du fonds de prévention du tabagisme par une contribution sociale sur le chiffre d'affaires des fournisseurs agréés de produits du tabac. Cette contribution fait peser un risque majeur sur l'activité des distributeurs, pour la plupart des petites et moyennes entreprises,

Le présent amendement vise ainsi à trouver une solution de compromis entre la lutte contre le tabagisme- financée ce fonds -et la pérennité de ces acteurs économiques en remplaçant cette taxe par une augmentation équivalente des droits de consommation spécifiques dont sont redevables les fabricants de tabac. intègre les dispositions de l'amendement n° 426 du Gouvernement relatif à la fiscalité des cigares et cigarillos et garantit ainsi l'atténuation de la hausse de la fiscalité, conformément à ses engagements auprès de la Confédération des buralistes.

cet amendement, dans le même esprit que celui qui vient d'être défendu par mon collègue Pierre Médevielle, vise à remplacer la taxe sur les fournisseurs de produits de tabac, créée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, par une augmentation des différentes composantes du droit de consommation sur le tabac.

Dès lors, en l'absence de répercussion de son coût sur les fabricants, les distributeurs se retrouveront dans l'impossibilité de payer cette taxe, qui s'avère ainsi confiscatoire. Troisièmement, la taxe fait peser un risque économique considérable sur la pérennité des distributeurs, qui sont souvent de petites et moyennes entreprises à la santé économique fragile, réparties sur l'ensemble du territoire. territoire. Quatrièmement, il existe de nombreux risques juridiques. Cette taxe suscite aujourd'hui une extrême tension dans l'ensemble de la filière, sachant que les solutions ne peuvent guère venir d'un cadre contractuel, dès lors que les obligations fiduciaires et légales des entreprises leur interdisent de payer des contributions dont elles ne sont pas les redevables légaux. Le remplacement de cette taxe par une augmentation, à due proportion, des droits de consommation spécifiques de l'ensemble des produits du tabac garantira des recettes fiscales équivalentes, assurant ainsi le financement des activités du fonds, tout en protégeant les distributeurs des conséquences économiques négatives de cette contribution. Ainsi, les recettes du fonds de prévention du tabagisme seront protégées, conformément aux objectifs de santé publique fixés par le Gouvernement. Je tiens également à préciser que la répartition entre part proportionnelle et part spécifique a été préservée afin de respecter la volonté gouvernementale de ne pas déséquilibrer les droits d'accise. Enfin, il convient de noter que cette disposition n'aura pas d'incidence sur les prix,

pour protéger les petits fournisseurs. Or il semblerait que la sécurité juridique de l'ensemble du dispositif ne soit pas assurée. Un autre pays européen qui avait mis en place une taxe identique a dû la retirer.

on ne peut réduire le nombre de fumeurs sans que l'activité de la filière diminue. Quand on veut vendre des armes, l'industrie de l'armement se développe ; quand on veut vendre des sucettes, l'industrie de la sucette se développe. Quand on veut moins vendre de tabac,

Pour au moins trois raisons, notre commission était opposée à la création de la taxe sur les fournisseurs agréés. Premièrement, les effets concrets de cette taxe sont difficiles à apprécier, car les relations commerciales entre fabricants et fournisseurs sont mal connues, en particulier les marges des uns et des autres. Deuxièmement, le produit de la taxe serait concentré sur quasiment un seul opérateur, Logista France, qui représente 98

il n'est pas opportun d'augmenter les dispositifs fiscaux déjà nombreux. L'effet recherché par cette taxe pourrait être atteint par une hausse des droits de consommation. nous pourrions être favorables à un dispositif supprimant la taxe sur les fournisseurs et augmentant à due concurrence les droits de consommation, à la condition que ce dispositif ne modifie pas la structure de la fiscalité et ne crée pas de distorsions entre les différents produits du tabac.

en en prévoyant la réévaluation annuelle. Notre commission s'est opposée au principe même de cette taxe, en particulier dans la mesure où l'objectif

vous le savez, les droits d'accise sont à la charge des consommateurs finaux, alors que la taxe créée l'année dernière correspondait à un objectif bien précis : mettre à contribution le secteur du tabac dans sa globalité, en partant du constat que les bénéfices réalisés sur les ventes de tabac, lorsqu'ils sont réalisés en France, échappent quasiment à tout impôt. Dès lors, il ne nous semblait pas pertinent de nous priver de cet outil fiscal qui joue un rôle différent de celui des accises dans le circuit allant de la production à la consommation.

Si nous partageons le même objectif final et la volonté de maintenir un fonds qui nous permette de lutter efficacement contre le tabagisme en France, nous devons être certains qu'il n'y ait pas de difficultés juridiques et organisationnelles. Or ce que vous proposez est complexe. En premier lieu, le rendement de la taxe n'est connu qu'en année n+1, au titre de l'année n. Il n'est donc pas possible d'ajuster le taux au 31 décembre. Si l'objet de l'amendement est bien de renvoyer l'ajustement du taux au pouvoir réglementaire, la disposition serait probablement contraire à la Constitution. Enfin, toujours au regard des règles constitutionnelles, il semble également risqué de prévoir que le taux puisse être fixé en fonction du rendement, sans considération aucune pour le risque que cette imposition soit confiscatoire en cas de forte baisse de la valeur du marché. en vous assurant de notre entière vigilance pour maintenir des ressources suffisantes et pour la prévention et pour le fonds, je préférerais que vous retiriez cet amendement ; à défaut, je

Je veux bien insister sur un point : l'amendement que j'ai défendu n'a nullement pour objectif de diminuer les prélèvements sur les ventes de tabac.

de manière équitable sur les fabricants de tabac, mais également de la sécuriser en évitant les nombreux contentieux liés aux difficultés de répercussion de la contribution par les distributeurs sur les fabricants.

Il est quand même particulièrement injuste que cette taxe repose exclusivement sur les distributeurs- ils en seront d'autant plus fragilisés -, même si nous sommes conscients qu'il faut trouver des fonds pour lutter contre le tabagisme. La parole est à M. le ministre. Nous n'allons

suivra l'avis du Gouvernement.

Cet amendement vise à instaurer une mission de suivi et d'évaluation des mesures d'augmentation du prix du tabac, afin de mesurer l'effectivité d'une telle décision en matière de santé publique et ses conséquences sur les buralistes. La consommation de tabac est une cause évitable de mortalité, puisqu'elle entraîne cancers et maladies cardio-pulmonaires.

Toutefois, il paraît souhaitable de procéder à l'évaluation de cette décision : évaluation de l'augmentation du prix du tabac et de la baisse espérée de la consommation ; évaluation des ventes parallèles, qui arrivent jusqu'en Corrèze, vous l'avez dit, monsieur le ministre

en matière notamment de santé publique. Nous l'avons dit hier soir, la corrélation entre la hausse des prix du tabac et la baisse du nombre de fumeurs n'est pas établie. Par ailleurs, les hausses successives mettent en difficulté les buralistes, qui comptent parmi les commerçants de proximité les plus importants, notamment dans les territoires ruraux et enclavés, par la diversité des offres qu'ils proposent. Quel est l'avis de la commission ? Le Gouvernement

la consommation de tabac en France. Monsieur Requier, le lien entre la hausse du prix du tabac et la diminution de la consommation de tabac a été prouvé dans tous les pays du monde, y compris dans le nôtre. En effet, le premier plan Cancer

des drogues et des toxicomanies est chargé, en lien avec le ministère de l'intérieur et du budget, de mesurer les ventes de tabac dans le réseau des buralistes et d'estimer le commerce illicite. Ces différentes données permettent de suivre à la fois la consommation et la vente de tabac en France. Même si les outils existants peuvent toujours être améliorés, il me semble qu'il n'y a pas lieu de confier au Conseil des prélèvements obligatoires une mission parallèle. Telle est la raison pour laquelle je suis défavorable à ces amendements.

La lutte contre le tabagisme, notamment par le biais de la fiscalité, ne fonctionnera pleinement que si, dans le même temps, les efforts sont concentrés sur la lutte contre la contrebande. Quel

dans le cadre de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016. Surtout, les services des douanes que nous avons auditionnés nous ont expliqué que le problème ne provenait pas tant du montant des sanctions que de leur application effective. À cet

de la commission ? La commission s'est interrogée sur cet amendement, qui vise à modifier l'un des échelons de la composante CO2 de la taxe sur les véhicules des sociétés.

comme cela existe déjà pour les véhicules fonctionnant au gaz naturel carburant ou au gaz de pétrole liquéfié. La parole

et les véhicules diesel. Cette convergence s'inscrit d'ailleurs dans la continuité des actions engagées par la France dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, ainsi que dans le développement des territoires à énergie positive pour la croissance verte, qui sont désormais plus de 400

sont des véhicules propres. Ce chiffre éclaire également le débat précédent, et étaye la nécessité d'adopter des mesures fiscales permettant enfin le développement des véhicules propres. Nous avons beaucoup trop de retard

et les entreprises et les salariés. Il vous est donc proposé, mes chers collègues, de neutraliser le surcoût lié à la différence de prix

la consommation de sucre, plus particulièrement sous forme liquide, a des conséquences lourdes sur la santé publique, notamment sur la santé des plus jeunes. Alors que les états généraux de l'alimentation sont ouverts, alors que l'on promeut une alimentaire saine, sûre, durable et accessible à tous, à l'heure où, dans le PLFSS, l'accent est mis sur la prévention, difficile de faire l'impasse sur ces boissons sucrées qui agrémentent notre quotidien. Loin de moi l'idée de faire un procès au sucre

pour atteindre le quota des 100 grammes journaliers au-dessus duquel vous mettez votre santé en danger. On comprend facilement le bouleversement engendré par ce type de breuvage chez les plus au sucre. Concrètement, en buvant deux verres par jour, votre poids augmentera de 400 grammes par mois. Inutile d'évoquer les effets sur les enfants, qui sont encore plus graves, puisque la prise de poids s'installe plus profondément ... Comme vous le savez, mes chers collègues, l'ensemble des boissons contenant une quantité même minime de sucres ajoutés sont taxées depuis 2013. La modulation de la taxe soda en fonction du taux de sucre dont il est question aujourd'hui prévoit que les boissons seront taxées de manière progressive en fonction du taux de sucre ajouté qu'elles contiennent. Cette taxe est donc juste, intelligente, intelligible, et elle évite les effets de seuil. Elle est incitative plutôt que coercitive pour l'industrie alimentaire- il est ici question d'éducation, non de répression. On comprend qu'elle ne vise pas à renflouer les caisses, mais qu'elle a pour objectif d'inciter fortement les industriels à diminuer la dose de sucre dans les boissons. Je salue aussi le courage de M. Véran, qui a pris en compte les réclamations des industriels qui regrettaient que certains produits avec édulcorants se retrouvent plus taxés que les produits avec sucres.

politiques de l'Assemblée nationale, visant un objectif de santé publique que nous partageons tous : limiter les risques d'apparition d'un certain nombre de maladies comme l'obésité ou le diabète de type 2, notamment chez les enfants.

Mme Pascale Gruny. Dans sa rédaction actuelle, l'article 13 prévoit une modification de la taxe sur les boissons avec sucres ajoutés, une progressivité étant instaurée en fonction de la quantité de sucres contenus, et une division par deux de l'actuelle taxe sur les boissons édulcorées.

hormis pour une partie de la population bien identifiée. En outre, cette modification de la taxe va amener les industriels,, à utiliser davantage d'édulcorants pour éviter de payer une taxe sur un sucre produit par une filière agricole qui est déjà confrontée à la fin des quotas de sucre.

et alors que les états généraux de l'alimentation sont toujours en cours, il apparaît important de poursuivre la concertation engagée par les acteurs de la filière - celle-ci vise à construire une politique équilibrée et efficace, reposant sur plusieurs leviers, fiscalité, prévention, éducation de reporter aux conclusions de cette concertation la modification de la fiscalité des boissons. Par conséquent, il est proposé de supprimer l'article 13 pour maintenir le dans l'attente des résultats de ladite concertation. Quel est l'avis

du Gouvernement ? La mesure proposée rend cumulables les taxes sur les boissons sucrées et celles sur les boissons édulcorées. Les boissons qui contiennent à la fois des sucres ajoutés et des édulcorants de synthèse

: des hausses modérées n'ont eu aucun impact sur la consommation. Il faut des hausses très fortes. Une taxation de quelques centimes sur des boissons sucrées peut-elle modifier les comportements et réduire la consommation de sucre ?

d'obésité ... L'obésité et la surcharge pondérale font partie des pathologies pointées du doigt par l'OMS dans les pays occidentaux, et pas seulement sont certes liées à des changements d'habitude alimentaire, exploités, au sens économique du mot, sans connotation péjorative, par ceux qui fabriquent des produits alimentaires.

le panier des personnes vivant dans les quartiers les plus difficiles ou dont les moyens économiques sont relativement faibles, il n'est pas prouvé qu'elles se dirigent vers les produits qui coûtent le moins cher,

applicable aux produits alimentaires de la grande distribution ou de certaines marques, vise à informer les consommateurs sur les taux respectifs de sucre de gras et à les orienter vers ce

le dispositif envisagé, afin que la taxation incite les industriels à réduire la teneur en sucre dans leurs boissons avec sucres ajoutés. Un lissage plus fin a été introduit en séance publique.

Des discussions complémentaires sur le niveau du barème pourraient donc intervenir dans le processus parlementaire. » Par cet amendement, nous proposons donc un barème visant à respecter cet engagement parlementaire et gouvernemental. Il s'agit de mettre en oeuvre une modulation visant non pas à augmenter le rendement de la taxe, mais à proposer un barème plus lisse. Cela permet de limiter les effets de seuil et de diminuer le niveau de taxation en fonction de l'effort fourni de baisse des teneurs en sucre. C'est beaucoup plus incitatif pour les fabricants

certains gardent leur formule d'origine mondiale et multiplient les produits à faible teneur en sucre ; d'autres fabricants diminuent régulièrement la teneur en sucre de leurs produits pour habituer les consommateurs sans

A-t-on déjà vu quelqu'un faire la fête avec du soja ? Il me semble que les boissons festives sont plutôt d'une autre nature ... Je le rappelle, le soja est un aliment de substitution qui est prescrit par les médecins pour les enfants ayant des allergies. Comme vous le savez, la densité nutritionnelle

rapporteur général. Cet amendement de la commission vise à compléter le dispositif adopté à l'Assemblée nationale. Il s'agit, en quelque sorte, du troisième pilier de la modification qui a été apportée à la fiscalité des boissons non alcooliques, afin d'encourager les consommateurs à se tourner davantage vers les boissons non sucrées. Par cohérence, en effet, il tend à supprimer le droit spécifique applicable aux autres boissons, dont le montant est 0,54 euro par hectolitre. La perte de recettes qui résulte de la suppression de cette taxe dont le rendement s'élevait, selon nos informations, à 79 millions d'euros en 2016, sera compensée par la hausse des recettes générées par les nouvelles modalités de taxation sur les boissons sucrées et édulcorées,

Le département de l'Aisne, que je représente, est le premier département de France producteur de betteraves sucrières. Le sucre y représente donc une richesse importante.

je voterai bien évidemment cet article, qui va dans le bon sens. Pour autant, madame la ministre, comme M. Daudigny, cette histoire de barème me trouble quelque peu.

La taxe existe déjà : elle avait été votée sous le gouvernement antérieur au gouvernement précédent. À l'époque, une distinction avait été faite entre les sodas

Alors que, en 2014, on a considéré le soja comme devant être exclu des boissons de type soda, je ne vois pas quel argument nouveau

existe des écarts de fiscalité entre l'Andorre et la France, mais il existe aussi des écarts de fiscalité absolument intolérables entre les cigarettes achetées en Corse et celles achetées sur le continent. J'aimerais que l'on ait la même cohérence sur tous les éléments de santé publique. Je mets aux voix

à la mise à disposition des patients en France des médicaments les plus innovants ; c'est un sujet, madame la ministre, que vous connaissez parfaitement. Nous disposons en France d'un dispositif ATU, ou autorisations

Ma crainte porte non pas sur le chiffre d'affaires des grands laboratoires, qui font des profits à deux chiffres, mais sur le fait que

M. le rapporteur général. Cet amendement vise à aménager le mécanisme de la clause de sauvegarde, afin de rendre comparables les assiettes prises en compte d'une année sur l'autre pour le calcul de la contribution due en application du taux Lv ou du taux Lh. L'année dernière, un amendement gouvernemental avait eu pour objet de faire porter ces taux sur l'évolution du chiffre d'affaires brut des entreprises, c'est-à-dire sans en retrancher les remises conventionnelles versées par les laboratoires dans le cadre des contrats passés avec le Comité Subsiste cependant le principe de la déduction des remises et contributions versées au titre de la contribution pour la détermination de l'assiette de l'année n-1. Il en résulte

le sénateur, les délais de remboursement et le fait que certains patients français pourraient subir des pertes de chance. Comme vous le savez, lorsqu'un médicament est innovant et en voie d'obtenir une autorisation européenne de mise sur le marché, il bénéficie en France d'une autorisation temporaire d'utilisation, une ATU, de cohorte, qui prend généralement effet six mois ou un an avant l'autorisation de mise sur le marché. Par conséquent, les patients français bénéficient d'un dispositif unique au monde, qui leur permet d'avoir accès à des médicaments innovants un an

Les médicaments innovants, qui généralement font partie de la liste en sus, sont vendus à l'hôpital et vont bénéficier d'une augmentation du taux Lh. Cela prouve bien que nous prenons en compte les innovations pour adapter notre balance entre les médicaments très innovants et ceux

du calcul de déclenchement les contributions versées en année n-1 au titre de la clause de sauvegarde, nous serions dans l'embarras. Nous avons un objectif très ambitieux en matière de maîtrise de la dépense des médicaments. La clause de sauvegarde n'a pour seul but que de sécuriser le respect de cet objectif fixé dans l'ONDAM et les économies prévues. Son application, pour être efficace, ne doit pas reprendre d'une année sur l'autre les éventuels dépassements, faute de quoi l'on

de l'assiette prise en compte pour la détermination de la contribution due au titre de la clause de sauvegarde. Il s'agit ainsi d'étendre aux biosimilaires l'exclusion existant déjà pour les médicaments génériques, afin de ne pas pénaliser la diffusion de ces produits par une taxation désincitative.

sociale pour 2017, à savoir à 2 %, au lieu des 3 % prévus dans le présent projet de loi. Nous avons bien noté les efforts du Gouvernement pour réduire le coût des médicaments, mais la marge financière reste tellement importante qu'il convient d'abaisser le taux de progression du chiffre d'affaires des industriels à partir duquel ceux-ci sont soumis à une contribution pour les médicaments distribués à l'hôpital. Certes, vous avez indiqué à l'Assemblée nationale, madame la ministre, que le relèvement de ce taux par rapport à l'an dernier était destiné à anticiper l'arrivée de nouveaux médicaments et de nouveaux traitements onéreux, notamment en cancérologie. néanmoins qu'un taux de 2 % n'empêche en rien l'innovation, tout en apportant des garanties plus solides quant à la maîtrise des prix. Je crois que chacun se souvient, ici, des dérives liées au Sovaldi pour la prise en charge de l'hépatite C. Ce médicament est le plus cher de l'histoire, alors à un coût très faible ! Je rappelle que la Cour des comptes a rendu en septembre dernier un rapport préconisant justement de mieux maîtriser le prix des médicaments. Elle recommandait, notamment, de donner plus de moyens au CEPS pour lui permettre de réviser plus régulièrement les prix des médicaments, en particulier pour les médicaments innovants et coûteux. Je souhaiterais, madame la ministre, que vous puissiez nous répondre sur ce point. Je sais que vous avez essayé d'oeuvrer dans ce domaine lors de lors de vos précédentes fonctions, notamment, mais il est important d'essayer de changer les règles en vigueur qui font qu'un pays comme la France n'a pas toute latitude pour fixer ses prix, le marché étant international.

issus tout au plus d'une vingtaine d'entreprises. Le taux de 3 % proposé permet de concilier la nécessaire prise en compte de l'innovation médicamenteuse, dont le retour constitue un motif de satisfaction,

à la fois grâce au taux élevé à 0 % et à la baisse de 50 % du prix des médicaments de la liste en sus, qui font l'objet de brevets anciens. Nous mettons la pression sur les mécanismes de rentes de situation ; le taux Lh nous permet simplement d'assurer l'avenir pour que les patients français accèdent à des innovations exceptionnelles.

La séance est suspendue.